La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à démocratiser le sport en France Mes chers collègues, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l'hémicycle, y compris pour les orateurs qui s'expriment à la tribune, conformément à la décision de la conférence des présidents, réunie le 1 décembre dernier. J'invite par ailleurs chacune et chacun à veiller au respect des gestes barrières.

ans jour pour jour, dans la nuit du 17 au 18 janvier 1998, je remportais en Australie le premier titre de championne du monde de natation d'une anniversaire vous confier ma fierté de présenter devant la représentation nationale du pays qui m'a accueillie à l'âge de 10 ans cette proposition de loi essentielle pour le sport. À deux ans des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, je souhaite que ce texte positionne le sport français en tête de file sur les questions d'éthique, de démocratie et d'intégrité. Cette compétition a nourri les rêves de beaucoup de mes nuits et l'ambition de nombre de mes jours. Elle porte en elle des perspectives d'éducation et d'émancipation, en particulier pour les femmes. Le monde du sport doit assumer cette ambition avec fierté et la France se doit de l'affirmer d'une voix claire et unie.

originale, allait droit au but : « démocratiser le sport en France ». Démocratiser le sport, c'est le rendre plus accessible à tous, sur tous les territoires, à tous les âges et les moments de nos vies. Démocratiser le sport, c'est aussi parler de transparence dans le fonctionnement des instances et la tenue des élections, c'est s'interroger sur la participation des femmes et des hommes aux décisions, c'est faire en sorte que toutes et tous puissent accéder à toutes les fonctions, y compris de présidence. messieurs les sénateurs, à vous aussi j'aimerais dire un grand merci, pour avoir oeuvré avec moi afin que cette proposition de loi trouve sa place ici, afin qu'elle puisse être enrichie de vos amendements et de ceux du Gouvernement, ainsi que de notre travail commun.

Ce satané virus nous a tous désarçonnés, mais il ne doit pas entraver notre volonté collective de progresser ! « Mieux faire ensemble », voilà le slogan qui a guidé mes premiers pas au ministère. Je l'aime, car il correspond à ma nature profonde. Il a permis en 2019 la création de l'Agence nationale du sport, opérateur de l'État doté d'un modèle innovant de gouvernance partagée au service du sport et de son développement.

Ma méthode pour y parvenir a été de considérer comment, au côté de l'État, chacun pourrait mieux y contribuer : les acteurs historiques du sport que sont le mouvement sportif et les collectivités territoriales, les parlementaires, évidemment, mais aussi le monde économique. Mieux faire ensemble », voilà aussi la devise qui a guidé la construction de ce texte ; je le dis sans présager de sa rédaction finale, car avoir grandi dans un pays totalitaire fait de moi une farouche défenseuse de l'expression démocratique.

ce point confiance aux athlètes et à leurs entraîneurs, car j'ai été moi aussi sportive de haut niveau et je sais à quoi ils pensent tous les jours. À deux ans de cette échéance, il est tout aussi important de renforcer la responsabilité sociale et environnementale du sport.

Vous le savez comme moi, le monde du sport est multiple ; s'il doit être au service de l'intérêt général, il faut veiller en permanence à ce que les intérêts particuliers ne l'emportent pas. C'est pourquoi je me suis réjouie que votre commission ait adopté un amendement tendant à compléter l'intitulé de cette pour préciser qu'elle vise à « améliorer la gouvernance des fédérations sportives ». J'ai un instant cru que nous allions partager cette vision moderne d'un sport conscient de la société dont il fait partie et du rôle crucial qu'il y joue

Je ne vous cache pas, monsieur le rapporteur, que j'aimerais ne pas seulement y croire : j'aimerais le faire ! J'aimerais que cet instant existe, au cours des deux jours et deux nuits que nous passerons ici ensemble. J'aimerais que nous soyons tous, instances sportives comprises, à la hauteur de ce que le sport représente dans la vie de nos concitoyens. un moment de progrès sensible, un instant suspendu où un regard bienveillant se pose sur vous pour vous dire : « Tu peux être encore meilleur demain ! » Être meilleur demain, c'est ce qui est attendu de nous tous, ici réunis. Le chemin de la modernité, du progrès et du courage est grand ouvert : il ne tient qu'à nous, qu'à vous, de l'emprunter. Oui, je suis très attachée à ce texte, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il lève des barrières et exprime l'ambition que le sport devienne une solution.

Le sport est un outil puissant pour la confiance en soi, pour l'autonomie et pour le bien-être des usagers, souvent fragiles, de ces établissements, notamment quand ces personnes sont en situation de handicap. C'est une avancée incontestable que

ancrer les savoirs sportifs fondamentaux, garantir trente minutes quotidiennes de sport à l'école : voilà autant d'avancées inédites. Tous ces dispositifs ne relèvent pas de la loi, mais ce débat me permettra de vous exposer la vision du Gouvernement et de rappeler l'action utile déjà concrètement déployée par Jean Michel Blanquer et moi-même pour révolutionner la place du sport à l'école, dès le plus jeune âge. Je veux à ce propos remercier ici tous les agents de notre grand ministère pour leur implication dans l'ensemble de nos politiques publiques proposition de loi est de permettre au monde sportif de prendre pleinement sa part dans des combats universels comme l'égalité entre les femmes et les hommes, ou encore la lutte contre toutes les formes de violence ou de discrimination. Nous avons déjà pleinement engagé le monde sportif dans la protection du pacte républicain, avec la loi confortant le respect des principes de la République ; il nous faut maintenant aller plus loin. Rénover en profondeur la gouvernance fédérale est un enjeu fondamental pour le sport français, mais aussi au-delà. Parce qu'il est pratiqué en club par 16 millions de personnes et regardé par l'immense majorité de nos concitoyens, le sport est une vitrine qui doit inspirer. Je veux donc assurer la parité au sein des instances dirigeantes des fédérations et de leurs ligues régionales. Je veux donner aux clubs une place plus centrale dans le mode de scrutin de l'élection des dirigeants. Je veux limiter le nombre de mandats des présidents et, demain, des présidentes. Enfin, je veux garantir l'honorabilité des acteurs sportifs, pour que des personnes condamnées pour violences sexuelles ne puissent pas entrer en contact

est le sens de l'histoire ; le mouvement sportif est prêt, il est disposé à engager sa révolution. Je vous invite donc, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, à ne pas manquer ce rendez-vous unique. Le titre III comprend enfin des dispositions essentielles pour renforcer et sécuriser le modèle économique du sport. Nous sommes encore plongés dans la crise sanitaire ; il faut donner au sport amateur et professionnel la possibilité d'en sortir le moins abîmé possible, tout en préservant notre modèle un ministère qui pilote et protège, et des fédérations qui exercent en responsabilité leur rôle en appui des ligues professionnelles qu'elles ont créées. Le Gouvernement a consacré près de 8 milliards d'euros au secteur sportif depuis le début de la crise. pour le secteur amateur et ses associations sportives, pour le sport professionnel, pour les loisirs marchands, ou encore pour le secteur de la montagne.

des violences discriminatoires et des violences physiques qui blessent et humilient. Ces violences doivent cesser ! Le Gouvernement défendra donc un amendement visant à créer une procédure d'amende forfaitaire en la matière, à la suite des engagements pris récemment avec le monde du football.

ce sens. Je me suis toujours engagée auprès de celles et de ceux qui font vivre le sport ; les supporters, les vrais, en font pleinement partie ! L'instance nationale du supportérisme doit nous permettre de mieux les écouter. Ainsi, le sport restera une fête,

La proposition de loi, examinée par les députés et adoptée au mois de mars 2021, était limitée dans ses objectifs, puisqu'elle visait essentiellement à réformer la gouvernance des fédérations sportives.

Grâce au travail du Sénat, la proposition de loi dont nous abordons la discussion aujourd'hui répond davantage aux enjeux auxquels doit faire face le sport français. Le développement du sport-santé, du sport en entreprise et du sport à l'école a été renforcé. Plusieurs mesures visant à mieux lutter contre les violences dans les stades ont été intégrées. Des amendements visant à allonger la durée du premier contrat professionnel de trois à cinq ans, deux amendements importants concernant la diffusion des compétions sportives, ainsi que des amendements tendant à entourer la reconversion des sportifs ont également été adoptés en commission.

Je pense au rôle du ministère des sports, qui est devenu incertain avec la création de l'Agence nationale du sport (ANS), à une meilleure répartition des missions entre les différents échelons de collectivités territoriales ... Tous ces sujets attendront le prochain quinquennat. Notre mission aujourd'hui est plus modeste, mais elle n'en est pas moins utile et importante. Nous pouvons trouver un accord pour faire aboutir un texte qui apportera des réponses à des problèmes urgents.

Le premier sujet a trait aux avancées à préserver concernant le sport-santé. Madame la ministre, nous partageons votre volonté de généraliser l'offre d'activités physiques et sportives dans les établissements médico-sociaux, mais nous ne nous faisons pas d'illusion : sans moyens dédiés, elle restera une simple déclaration d'intention. Aussi attendons-nous des engagements financiers de votre part, lesquels conditionneront le rétablissement du dispositif du référent.

Elle est maintenant renvoyée à un autre débat. L'extension du dispositif à de nouveaux publics constitue une avancée certaine. Nous avons néanmoins tenu à mieux l'encadrer pour la rendre réellement opérationnelle, dans le cadre du parcours de soins coordonné. La commission a également souhaité formaliser l'existence et les missions des maisons sport-santé dans le texte, car, sans véritable structuration de la filière, le sport sur ordonnance ne pourra pas se déployer à une plus grande échelle. deuxième sujet porte sur l'accès aux équipements sportifs scolaires, qui ne peut se faire à n'importe quel prix pour les collectivités territoriales. De nombreux établissements scolaires disposent d'équipements sportifs Je partage l'idée de faciliter leur utilisation par des associations et clubs sportifs, des établissements de l'enseignement supérieur ou des entreprises en dehors du temps scolaire : le soir, le week-end ou encore pendant les vacances scolaires. En cela, l'aménagement d'un accès indépendant aux équipements sportifs lors de la construction d'un nouvel établissement scolaire est une mesure importante. D'ailleurs, de nombreuses collectivités n'ont pas attendu ce texte pour mener cette réflexion et prévoir cet aménagement dans les plans de construction de la nouvelle école, du nouveau collège ou du nouveau lycée. En revanche, l'obligation, sans exception possible, d'aménager un tel accès, en cas de travaux importants de rénovation, risque d'être contre-productive. En effet, certaines collectivités pourraient renoncer à rénover leurs équipements sportifs scolaires accès indépendant ou au coût trop élevé de cette opération. C'est pourquoi il a semblé important à la commission d'introduire un assouplissement à cette obligation : le coût de ces travaux d'aménagement par rapport au coût total de rénovation doit être pris en compte.

Nous sommes tous conscients de la nécessité de faire évoluer cette gouvernance. Toutes les fédérations sportives sont confrontées à de nouveaux enjeux. La pratique sportive évolue, des investissements sont nécessaires. La politique en faveur des sportifs de haut niveau n'a pas encore trouvé son équilibre. Pour mener à bien ces chantiers, les fédérations doivent attirer de nouveaux profils, plus jeunes, plus entrepreneurs, plus féminins, plus internationaux dans leur approche. Nous partageons donc votre ambition d'accompagner le renouvellement des dirigeants, mais celui-ci ne peut être imposé contre le mouvement sportif, en faisant fi de la réalité de la situation des fédérations. Ces dernières ont renouvelé leurs dirigeants au printemps dernier. De nouveaux présidents ont été élus, qui sont parfois des présidentes.

qui a permis d'établir qu'il n'y avait pas d'accord pour que les évolutions nécessaires soient imposées par le haut, c'est-à-dire par la loi, de manière autoritaire. Je crois qu'il faut entendre ce message et faire davantage confiance aux dirigeants du mouvement sportif. C'est le sens des amendements qui ont été adoptés en commission. Oui à la parité intégrale quand elle est possible ! Donnons-nous seulement encore un peu de temps pour former les dirigeantes là où c'est nécessaire. Oui à plus de démocratie dans le processus électoral, en donnant une place primordiale aux clubs, mais sans distinguer selon leur forme, pour tenir compte de la diversité d'organisation des fédérations. Oui, enfin, au renouvellement des présidents, mais sans imposer des limitations qui n'existent pour aucun autre type d'associations. Sur ces trois sujets, les propositions que nous formulons constituent un compromis crédible et réaliste entre votre ambition et le respect de l'autonomie du mouvement sportif. Le quatrième sujet porte sur les garanties indispensables pour permettre d'accompagner le redressement du football professionnel.

dramatique que connaît le football français- j'allais dire « désespérée », mais elle ne l'est pas tout à fait justement, puisque la ligue a travaillé sur plusieurs projets pour redresser la barre et rétablir l'attractivité de sa compétition phare. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous : nous sommes attachés à notre modèle français qui délègue aux ligues professionnelles l'organisation et la gestion du sport professionnel. Nous n'envisageons pas de revenir sur cette répartition des rôles. L'amendement adopté en commission permet de rappeler des principes et d'affirmer des valeurs. Dans notre modèle, c'est la fédération sportive qui doit rester garante de l'intérêt général et de l'avenir de la discipline, chacun aujourd'hui en convient. Le dialogue rétabli entre la fédération et la ligue a permis de réaffirmer cette évidence. C'est pourquoi j'ai décidé de proposer en séance une nouvelle rédaction de l'article 10 A, qui tire les conséquences de nos échanges avec la fédération et la ligue. Cette nouvelle rédaction réaffirme le rôle de la fédération et prévoit sa participation dans les instances de la société commerciale ; en contrepartie, elle laisse la ligue assurer le fonctionnement de cette société. Cette nouvelle rédaction nous semble équilibrée et nous serons vigilants à ce que cela reste ainsi. En conclusion, mes chers collègues, je pense que l'ensemble des sénateurs, toutes sensibilités politiques confondues,

D'ailleurs, je rappelle que l'objectif était de voir trois millions de licenciés supplémentaires d'ici à 2024. C'est dans ce contexte, renforcé d'ailleurs par un contexte de crise sanitaire mondiale, que ce texte nous est présenté. Pourtant, le 20 décembre 2017, devant l'Assemblée nationale, la ministre des sports d'alors, Laura Flessel, déclarait souhaiter présenter au début de 2019 devant le Parlement un projet de loi Sport et société, visant à encourager la pratique pour tous et partout, tout au long de la vie. Malheureusement, nous avons dû attendre jusqu'à ce 18 janvier 2022 pour qu'un texte nous arrive en séance publique. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais

Premièrement, sans pour autant répondre au manque d'encadrants dans les associations sportives, le texte permet de libérer des espaces pour la pratique libre. Notre groupe ne peut que partager cet objectif, tant on sait à quel point le sport peut s'apparenter à une oxygénation. Combien de fois avons-nous vu des jeunes escalader la grille des écoles pour jouer au foot ou au basket dans la cour le week-end ? Tant de fois que certaines mairies laissent aujourd'hui les portails ouverts ! Les dispositions du texte permettent tout à la fois de sécuriser les pratiquants, mais aussi les écoles et les collectivités territoriales.

entre les femmes et les hommes a permis quelques avancées, il faut aujourd'hui aller plus loin. Ce texte nous permet de dégager un horizon, dans un calendrier par ailleurs tenable. maintenant aux limites que nous voyons à ce texte. Se pose bien évidemment la question du coût. Selon une étude de 2018, près de 57 % des Français considéraient que le prix des licences et des équipements était le principal frein à leur pratique. J'étais d'ailleurs samedi après-midi avec les jeunes de l'Espace Jeunes municipal de Septèmes-les-Vallons, commune située au nord de Marseille, qui me faisaient justement remarquer que, dans un texte visant à la démocratisation du sport, pas un mot sur le prix des licences, pas un mot sur le coût pour suivre le sport à la télévision, pas un mot non plus sur le coût pour assister à de grands événements sportifs. Ainsi, alors que la majorité des épreuves des jeux Olympiques de 2024 auront lieu en Seine-Saint-Denis, combien de jeunes issus des quartiers populaires de ce département pourront matériellement assister à ces épreuves, s'ils le désirent ? Très bien ! Nous sommes donc bien loin de la grande loi de démocratisation attendue. Parmi les leviers qui nous semblent sous-exploités se trouve la question de la visibilité. il faut le rappeler, il existe un lien très clair entre la médiatisation d'une discipline et sa pratique. On peut ainsi citer le triplement des licenciés en canoë-kayak, handball et natation, consécutif à un dispositif de médiatisation favorisé par des générations dorées. Or on ne peut que s'inquiéter de la disparition progressive du sport diffusé en clair, toutes disciplines cumulées. C'est d'autant plus regrettable que, à nos yeux, la démocratisation de la pratique ne peut que se faire en parallèle d'une démocratisation de la diffusion et de la gouvernance. Se poursuit par ailleurs une forme d'hypocrisie dans notre conception du sport. Pratique populaire, à tous les sens du terme, on valorise dans la communication l'ambiance des stades et les moments de communion. Ainsi, dans son clip promotionnel, la Ligue de football professionnel (LFP) utilise des images des stades avec une multitude de fumigènes, car elle sait bien que cela est vendeur

Reste enfin la question de la société commerciale, que la LFP est en train de monter en parallèle de nos discussions. On l'a bien compris, son seul intérêt aujourd'hui est d'injecter de la trésorerie en urgence, après l'échec et le scandale de Mediapro. À son sujet se posent encore de multiples questions. Quelle capitalisation et quelles retombées économiques à long terme ? Quelle clé de répartition entre le monde amateur et le monde professionnel et au sein même des clubs professionnels de ligue 1 ? Quelle base de calcul pour le décider ? Autant de questions auxquelles nous aurions aimé avoir des réponses avant l'examen de ce texte. Cela revient

et n'a pas su enrayer l'inquiétude née de la crise traversée par le sport amateur. Où est passée la grande loi Sport et société qui devait ancrer une approche ambitieuse de la politique sportive de demain, cette grande loi qui devait faire du sport une grande cause nationale, permettre d'augmenter le nombre de pratiquants, d'oeuvrer en approche fine des territoires, de simplifier, de traiter enfin du bénévolat Autant de sujets sur lesquels nous ne manquons pas d'interroger et de bousculer régulièrement le Gouvernement et qui, malgré tout, restent largement en suspens ... Ce texte aurait dû constituer la base d'un projet de loi attendu en 2019 ou 2020. À défaut de pouvoir déposer un tel texte en bonne et due forme, madame la ministre, vous avez décidé à l'été 2020 de susciter cette proposition de loi. Cette méthode présente en l'espèce, comme vous le savez, plusieurs inconvénients.

la plupart des dispositions correspondent à des ajustements et ne traduisent pas une vision renouvelée de la place du sport dans la société : on voit mal comment les dispositions prévues pourraient contribuer de manière effective à amener à la pratique sportive les populations qui en sont éloignées. De même, l'effectivité de la mise en oeuvre opérationnelle des projets sportifs territoriaux, dispositions de nature administrative, reste largement dépendante de la capacité des collectivités locales à dépasser leurs divisions, malgré la lourdeur du dispositif. la ministre, faute d'être adossées à un volet financier solide et sans garanties de votre part, plusieurs mesures ont malheureusement une portée plus déclarative qu'opérationnelle. Je pense au dispositif du « référent sport » que la commission n'a pu valider en l'état, mais aussi à l'élargissement du sport sur ordonnance que la commission a dû retravailler pour permettre son maintien et faciliter son développement dans le cadre du parcours de soins coordonné. On le voit, et nous le rappelons régulièrement lors de l'examen des projets de loi de finances, le sport reste malheureusement le parent pauvre des politiques publiques. la ministre, nous ne pouvons que déplorer la pusillanimité avec laquelle le Gouvernement traite certains sujets, alors que la crise sanitaire qui se prolonge et dont on n'entrevoit guère l'issue aurait nécessité un signal fort financement des associations pourtant en grande souffrance et pour lequel vous renvoyez au Pass'Sport, mais aussi fonctionnement fédéral relégué à sa portion la plus congrue. Plus grave, certains autres sujets pourtant cruciaux, comme le bénévolat, qui nécessite accompagnement et valorisation, sont restés aux abonnés absents ! Concernant Concernant le développement de la pratique pour le plus grand nombre, on est donc loin de l'audace de la proposition de loi de 2019, qui prévoyait la création du « 1 % sportif », sur le modèle du 1 % culturel, qui aurait obligé tout maître d'ouvrage public à intégrer un équipement sportif à toute nouvelle construction, ou qui envisageait de relever le plafond des taxes affectées à l'Agence nationale du sport, laquelle distribue une large partie de son budget aux associations sportives.

un cadre d'organisation renouvelé, un accès aux équipements sportifs objectif et une vision des projets sportifs territoriaux affinée, au travers d'une approche pragmatique. Il a également permis d'enrichir le texte de dispositions visant à développer le sport à l'école, à mieux concilier études et pratique du sport de haut niveau ou encore à mieux valoriser l'engagement sportif à l'université. Je ne saurais oublier de mentionner des points plus particuliers sur lesquels nous avons travaillé et qui nous paraissent mériter votre adhésion, madame la sur certains d'entre eux, à savoir sécuriser la possibilité pour les ligues professionnelles de créer une société commerciale, garantir un renouvellement dans les fédérations sportives sans les déstabiliser ni s'ingérer dans leur vie démocratique, encadrer objectivement le supportérisme, permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de renouveler et d'adapter les primo-prescriptions d'activité physique adaptée (APA) effectuées par les médecins,

! Faites confiance aux dirigeants pour une bonne répartition dans les tribunes en respectant les mesures sanitaires. Croyez-moi : en faisant cela, vous vous ferez plein d'amis.

janvier 1998. Pour beaucoup de nos concitoyens, accéder au sport relève de la course d'obstacles, les barrières étant le plus souvent sociales ou territoriales. Il existe dans notre pays une véritable fracture sportive. Selon l'auteur du texte que nous examinons aujourd'hui, près de 42 % de la population ne pratique aucune activité physique. Ce chiffre pourrait s'aggraver avec le développement croissant de l'usage par les jeunes des écrans numériques, habitude qui, hélas ! les conduit de plus en plus à s'installer dans la sédentarité. Dans ces conditions, il reste beaucoup à faire pour encourager la pratique sportive de tous. C'était l'objet du texte : démocratiser le sport. Je dis bien « c'était », car, en raison des dizaines d'articles qui se sont greffés à la proposition de loi initiale, cet objectif s'est quelque peu dilué dans un ensemble de dispositions hétéroclites.

Quelle est au fond la problématique fondamentale dans l'accès au sport ? Si l'on s'en tient au sens strictement étymologique, l'accès au sport, c'est tout d'abord la possibilité de s'y rendre physiquement. L'offre sportive et son corollaire, la densité des équipements et des associations sportives, sont à l'évidence des facteurs déterminants. Si des stades de foot ne s'étaient pas installés au pied des immeubles, aurions-nous connu les Zidane, Matuidi et Pogba ? Sur ce volet, le texte apporte une réponse phare : l'ouverture des moyens sportifs scolaires et universitaires aux personnes extérieures. C'est un dispositif très intéressant qui joue la carte de la proximité. pour autant s'inquiéter des contraintes que cela pourrait induire en termes de responsabilité, d'organisation et de coût financier pour les collectivités locales ? Rappelons que celles-ci apportent déjà chaque année près de 12 milliards d'euros au financement des équipements sportifs et des associations sportives. L'accès au sport, c'est aussi un enjeu social que le texte ne prétend pas résoudre directement, même si l'ouverture à plus d'équipements devrait apporter des améliorations en la matière, ainsi que l'accent porté sur l'école au travers de plusieurs articles. La discussion budgétaire sur la mission « Sport, jeunesse et vie associative » que nous n'avons malheureusement pas eue au Sénat aurait permis de rappeler que les politiques publiques ont cette première mission d'inclusion de tous les publics, sans quoi l'objectif de cohésion sociale ne pourra jamais être totalement atteint. Comme le souligne le dernier rapport du Conseil d'État sur le sport, il est « souhaitable de recenser, soutenir et étendre les actions innovantes utilisant le sport à des fins d'insertion et d'émancipation Toute politique d'aménagement devrait promouvoir un urbanisme favorable à l'activité sportive et physique. Il faut développer les sites de plein air, les parcours sécurisés de marche et de vélo, multiplier les ou toutes sortes d'installations gratuites. Dans cet esprit, madame la ministre, le Pass'Sport est également une bonne initiative. Il faudra cependant l'évaluer pour s'assurer qu'il atteint ses objectifs, notamment auprès des ménages modestes. J'en viens au deuxième grand enjeu du texte, l'appui au sport-santé. À cet égard, la proposition de loi apporte des mesures bienvenues, par exemple l'inscription de l'offre d'activités physiques et sportives au titre des missions des établissements et services On peut toutefois s'inquiéter de la situation financière de certaines de ces structures, qui risque de compromettre son effectivité sur tout le territoire. Mon groupe regarde également avec intérêt la mesure d'élargissement du périmètre des prescripteurs de l'activité physique adaptée et l'extension du champ de ses bénéficiaires. Les bienfaits thérapeutiques du sport ne sont plus à démontrer. Il faut par conséquent encourager ce dispositif et, bien sûr, réfléchir à son modèle économique, car son absence de prise en charge par l'assurance maladie pose question. Si l'on considère que le sport est un médicament, ce dont je suis pour ma part convaincu, alors les financements doivent être à la hauteur. En effet, les gains pour la santé physique et psychologique sont immenses et les coûts évités le sont tout autant. En outre, cet élargissement doit s'accompagner du développement de la formation à l'encadrement de personnes qui présentent des pathologies chroniques ou des limitations fonctionnelles. Les modules de formation Activité physique adaptée, dispensés au sein des instituts nationaux supérieurs du professorat et viens aux articles intéressant la gouvernance des fédérations sportives. Tout ce qui peut inviter ces instances à se régénérer et se féminiser va dans le bon sens, celui d'un monde sportif ouvert et conforme aux valeurs d'égalité et de fraternité qui lui sont théoriquement consubstantielles. Attaché aux bienfaits du sport pour la santé et la cohésion sociale, le groupe du RDSE votera en faveur de cette proposition de loi. Compte tenu des nombreux apports qu'elle contient, ses membres souhaitent la voir adoptée définitivement dans les prochains mois et espèrent que la suspension des travaux parlementaires n'y fera pas obstacle. La parole

À mes yeux, ce texte aurait dû débuter par l'actualisation de la relation qui unit l'État et le mouvement sportif, c'est-à-dire la délégation pour mission de service public, toile de fond de cette proposition de loi. Le choix d'intégrer cette actualisation dans la loi confortant le respect des principes de la République, texte déjà examiné, relève quasiment de l'anomalie. de loi vise un objectif bien légitime : la démocratisation du sport, c'est-à-dire un développement du nombre de pratiquants, par la levée des obstacles qui entravent l'accès aux différentes Cette intention est louable, pour des raisons historiques- le fait sportif n'est pas encore véritablement reconnu pour son importance sociétale -, mais aussi pour des motifs conjoncturels. selon l'enquête de l'institut Ipsos, rendue publique à la fin du mois de décembre dernier, 66 % des sondés ont déclaré pratiquer un sport en 2021, contre 81 % en 2020.

nous appellerons à une plus grande démocratisation et à une plus forte territorialisation, non seulement des pratiques, mais également des organisations et des fonctionnements, dans le respect des débats menés récemment par le CNOSF, qui fédère l'ensemble des disciplines sportives, olympiques ou non, de notre pays.

Mettons-nous au diapason des jeux Olympiques de Paris : pour la première fois, nous aurons en 2024 des jeux paritaires. Mettons-nous au diapason du combat mené par Alice Milliat, cette sportive française qui avait su fédérer le mouvement sportif féminin en France puis au niveau mondial.

Un sujet a défrayé la chronique : la possibilité donnée à une ligue sportive professionnelle de créer une société commerciale chargée d'optimiser ses droits audiovisuels dès lors que la fédération concernée lui a transféré la responsabilité juridique de la commercialisation et de

Mais reconnaissons que les progrès relatifs à l'éthique du sport demeurent modestes, alors que, pour ne prendre qu'un seul exemple, selon la direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) des clubs, 60 % des agents de footballeurs échappent à toute réglementation.

Notre commission a déjà fait évoluer le texte de cette proposition de loi, souvent à partir d'amendements communs ou très voisins, par-delà nos sensibilités politiques. Nous continuerons à intervenir dans cet état d'esprit. Si nous voulons un pays plus juste et plus solidaire, il faut en passer par des réformes permettant d'acquérir de nouveaux droits et de nouvelles libertés.

à commencer par la solidarité, la fraternité, mais également le respect de l'engagement. En ces temps où la crise sanitaire a perturbé la pratique sportive de nos concitoyens, la majorité présidentielle s'est justement engagée pour le sport. Des dispositifs inédits ont été imaginés, notamment pour la jeunesse. De toute évidence, le Pass'Sport, que je ne cesse de promouvoir sur le terrain, est un succès. Mais il nous faut aller plus loin, pour encourager la pratique sportive. loi, tous les parlementaires, de l'Assemblée nationale comme du Sénat, de la majorité comme des oppositions, soient eux aussi engagés pour le sport et sa démocratisation en France. Son texte compte

D'abord, pour démocratiser le sport, nous devons toutes et tous encourager la pratique sportive. La France est une nation où le sport occupe encore une place singulière. Qu'il s'agisse des jeux Olympiques ou des grandes compétitions internationales, la France se démarque et, bien souvent, pour notre plus grand plaisir, la France gagne. Cependant, depuis le début de la crise, on observe une réduction de la pratique sportive dans le monde amateur, et une majorité d'acteurs éducatifs et sportifs soulignent l'urgence du renouvellement de l'offre sportive. Face à ce constat, les parlementaires que nous sommes doivent agir pour simplifier les procédures et supprimer les barrières inutiles. À titre d'exemple, les associations sportives auront auront désormais l'autorisation d'utiliser les équipements sportifs des collèges et des lycées, dans l'intérêt du plus grand nombre. La pratique sportive doit être l'affaire de tous. Nous devons donc l'encourager, y compris dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Démocratiser le sport, c'est aussi réformer la gouvernance des fédérations sportives dans notre pays. Sans faire le jeu des dogmes sectaires ou entrer dans les querelles de chapelle, je le dis sans ambiguïté : nos fédérations sportives doivent se remettre en question, qu'il s'agisse de parité, d'éthique ou encore d'intégrité morale. Un constat doit nous alarmer : les femmes ne sont pas assez représentées dans les instances des fédérations sportives. Les choses sont en train de changer, et c'est tant mieux.

à l'exigence de parité, la volonté du Gouvernement est d'agir pour changer les mentalités. En matière d'éthique, les fédérations sportives doivent être plus exemplaires et plus transparentes. Il nous faut modifier certaines règles. C'est ainsi que l'article 7 de la le nombre de mandats pouvant être exercés par les présidents de fédération. Je regrette sa suppression pure et simple, souhaitée par le rapporteur. Au nom de mon groupe, je voterai donc l'amendement du Gouvernement qui rétablit cet article 7 dans sa rédaction initiale. Le renouvellement régulier des instances fédérales, y compris régionales, est une condition indispensable au dynamisme des fédérations. C'est aussi la garantie du débat démocratique dans le monde sportif. Enfin, pour démocratiser le sport, encore faut-il renforcer le modèle économique sportif en général. Une fois encore, il est question d'exemplarité. Le texte propose l'ouverture des sociétés sportives à l'économie sociale et solidaire, mais aussi l'ajout de la société coopérative d'intérêt collectif à la liste des types de sociétés autorisés par la loi. Ce sont des mesures positives, mais peut-être insuffisantes. L'exemplarité est un levier parmi d'autres.

Mes chers collègues, le sport est un ensemble de valeurs, parmi lesquelles figure le respect. Qui de mieux que les arbitres pour garantir le respect sur le terrain ? Ces acteurs demandent une meilleure reconnaissance et une plus grande représentativité dans le monde sportif. Sur ce point, je salue l'amendement sur le statut des arbitres- ayant été moi-même arbitre -et des juges de haut niveau du sport professionnel. À titre personnel, je crois que nous devons aller encore plus loin pour garantir leur présence au sein des instances dirigeantes des fédérations sportives. La sécurité et le bien-être du public sont indispensables si l'on veut préserver la bonne santé économique du sport. En même temps, les mesures privatives de liberté et les sanctions ne doivent pas être disproportionnées. Il nous faut donc réformer les procédures, pour les supporters comme pour l'administration, et, surtout, favoriser la concertation entre les autorités publiques et les clubs. C'est dans cet état d'esprit que je défendrai un certain nombre d'amendements à propos des interdictions de stade administratives, commerciales et collectives. Je sais, madame la ministre, que vous êtes pleinement préoccupée par ces sujets. Je peux vous assurer de mon soutien et de ma volonté de travailler, dans l'intérêt des Français, pour un monde sportif plus respectueux.

Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour triompher, et la difficulté pour la vaincre. » Fondateur des jeux Olympiques modernes, il a été le premier à oeuvrer pour démocratiser le sport en France. L'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est une formidable occasion de renouveler cette volonté, et de placer le sport au centre de la vie des Français. Forger l'esprit d'équipe, donner le meilleur de soi-même, former à la loyauté et au fair-play : le sport véhicule des valeurs très fortes, et il favorise l'insertion sociale et l'épanouissement personnel. C'est une école de la vie et un élément essentiel pour souder les liens entre nos concitoyens. Au-delà de ses valeurs intrinsèques, le sport a de nombreuses vertus. L'activité physique adaptée est un levier essentiel de santé publique, agissant à la fois sur la prévention et sur la guérison.

étendre les prescriptions d'activité physique adaptée aux personnes atteintes d'une maladie chronique. Je pense que nous devons ouvrir ce dispositif au plus grand nombre possible de personnes dont l'état de santé nécessiterait la pratique d'une activité physique. physique. Je proposerai donc plusieurs amendements pour inclure dans le dispositif les personnes atteintes de troubles mentaux et les seniors en situation de dépendance, afin de limiter l'aggravation de leur perte d'autonomie. Pour donner une réelle portée au sport-santé, il appartient désormais au Gouvernement de généraliser la prise en charge des séances par l'assurance maladie. Certaines villes et certaines mutuelles le font déjà. Si le sport améliore l'état de santé général, il favorise aussi l'apprentissage, la concentration et la mémorisation. Le développement du sport à l'école est une priorité nationale. Nous devons, autant que possible, faciliter les liens entre les associations sportives locales et les établissements scolaires, et définir une stratégie nationale du sport à l'école et à l'université. La commission a adopté un amendement pour prévoir un temps minimal de pratique sportive quotidienne dans les écoles primaires. C'est un premier pas, mais nous devons être plus ambitieux. Jean-Pierre Decool et moi-même avions déposé des amendements pour étendre la pratique sportive quotidienne aux collèges, lycées et universités. Ces amendements ont été déclarés irrecevables, c'est regrettable. Pour encourager l'éducation sportive, nous souhaitons mettre en place à chaque rentrée scolaire une journée de découverte des sports, en partenariat avec les associations et les élus locaux. Cette journée, inspirée du modèle allemand, pourrait avoir lieu dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire, qu'il faudrait étendre aux universités. Enfin, je défendrai un amendement qui me paraît essentiel pour développer le sport en entreprise.

Dans cet objectif, je propose la mise en place d'un ticket sport, sur le modèle du ticket restaurant, pour permettre aux salariés de financer tout ou partie d'un abonnement à une pratique sportive. Actuellement, seulement 7 % des entreprises mettent à disposition de leurs salariés une offre sportive. La sédentarité est une bombe à retardement. Les professionnels de santé sont de plus en plus nombreux à nous alerter : un adulte sur deux ne pratique aucune activité physique, et les enfants passent de plus en plus de temps devant leurs écrans. Nous devons inviter le sport dans le quotidien des Français et atteindre l'objectif de trente minutes d'activité quotidienne. À mon sens, le sport-santé, le sport scolaire et le sport en entreprise sont les trois priorités pour démocratiser le sport en France.

pour voir enfin arriver ce texte au Parlement. Celui-ci avait pourtant été promis dès le début de ce quinquennat. Il vise à promouvoir la pratique du sport dans notre pays, donnant ainsi l'élan nécessaire à une nation qui, justement, doit accueillir les jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. C'est bien tard, et bien décevant. Sur la forme, à l'image d'un gruppetto lors d'une étape du Tour de France, ce texte est hors délai, et il faudra compter sur l'indulgence des commissaires de course que nous sommes pour un éventuel rattrapage. Sur le fond, cette proposition de loi comportait une succession de gestes sportifs mal maîtrisés, voire d'infractions aux règles sportives applicables sur tous les terrains de jeu. Je salue donc le travail considérable de notre rapporteur Michel Savin et de la commission, qui a permis d'enrichir ce texte.

Le rapport du Gouvernement introduit en commission nous éclairera sans doute utilement sur le sujet. Cela continue, avec une mêlée ouverte inorganisée dans l'article 1 et son chapelet de bons sentiments venant alourdir un code du sport qui mériterait tellement mieux. Dans ce même article, nous ne sommes pas loin d'un grossier passage en force, avec l'introduction surprenante de l'identité de genre : ces considérations inutiles ont judicieusement été supprimées en commission. Plusieurs hors-jeux ont été identifiés par de nouvelles obligations faites aux collectivités locales, évidemment sans compensation financière. Carton rouge ! J'en veux pour preuve les contraintes liées à la construction de nouveaux équipements sportifs ou à l'élaboration de plans sportifs locaux. Les intentions sont louables, mais leur concrétisation nécessite un geste budgétaire de la part de l'État. Il y avait aussi un refus de jeu manifeste, caractérisé par l'absence totale de considérations sur l'enseignement supérieur. Pourtant, après une scolarité bien encadrée par des horaires et des programmes nationaux, beaucoup d'étudiants cessent toute activité physique à l'entrée dans le supérieur, à un moment où cela constitue pourtant un élément essentiel J'ai proposé et fait adopter en commission plusieurs amendements visant à mettre à disposition des étudiants les équipements sportifs situés dans environnement proche. D'autres dispositifs plus ambitieux, comme celui réservant une demi-journée à la pratique du sport, mériteraient d'être examinés, même s'ils touchent à l'autonomie des universités. Puis, il y a ce jeu dangereux, qui consiste à masquer la réalité des choses et à ne surtout pas aborder les sujets délicats. Pourtant, les discussions sur le projet de loi le respect des principes de la République ont mis en lumière l'entrisme de certaines idéologies dans nos clubs de sport ainsi que dans nos établissements scolaires et universitaires. Nous le savons : le sport est un vecteur privilégié, et désormais bien identifié, pour atteindre et formater notre jeunesse. Notre responsabilité est de ne pas céder, et d'exiger la neutralité de chacun lors des compétitions sportives. Au nom du groupe Les Républicains, je vous proposerai un amendement en ce sens. Enfin, j'hésite entre le retour en zone et la passe en avant en ce qui concerne les dispositions liées à la gouvernance des fédérations sportives, dans un contexte particulier, lié à une crise sanitaire qui les a grandement fragilisées. extrêmement réservé, à titre personnel, sur l'imposition de quotas de toutes sortes dans notre société, et je considère que les nouvelles exigences de parité sont excessives et ne prennent pas assez en compte le mouvement engagé dans la très grande majorité des fédérations. Malgré tout, le Sénat s'est emparé sérieusement de ce texte, et je ne doute pas que nous poursuivrons en séance le travail de qualité engagé en commission. Espérons que le Gouvernement y sera attentif ne pratiquera pas un plaquage haut de mauvais aloi ! La parole

Après une si longue attente, nous aurions aimé obtenir un texte ambitieux et transversal qui redynamise la pratique de l'activité physique et permette l'avènement d'une société sportive ouverte et accessible à toutes et tous

Mais, à la lecture de cette proposition de loi, nous sommes relativement déçus. Comme beaucoup de textes de cette fin de mandat, celle-ci contient un catalogue de mesures, souvent utiles, certes, voire nécessaires. Mais la vision d'ensemble, le nouveau souffle pour une France sportive ne sont pas au rendez-vous. Il faut reconnaître que ce texte comporte des mesures qui, si elles ne sont pas révolutionnaires, méritent globalement d'être saluées. Je pense ainsi à l'ouverture de l'accès aux équipements sportifs des collèges et lycées pour les clubs, les étudiants et les associations, ou encore à l'établissement de plans sportifs locaux, qui permettront un meilleur accès à la pratique sportive en la démultipliant sur nos territoires. Je pense également aux mesures concernant l'honorabilité des instances dirigeantes des fédérations, au non-cumul des mandats dans le temps pour les présidents de fédérations, et à l'instauration d'une plus grande parité, même si ces deux dernières mesures ont été largement amoindries par notre commission. Saluons, enfin, la régulation du sport professionnel, avec la lutte conte la dérive des paris sportifs.

tout n'est pas à jeter dans l'apport du Sénat jusqu'ici, force est de constater que sa contribution aux mesures phares du texte ne va clairement pas dans le bon sens. Nous avons déjà entendu ces arguments, lorsque nous débattions de parité en politique : « Pas trop vite, les institutions ne sont pas prêtes, nous allons décourager des vocations Nous examinons donc un texte limité, et encore amoindri par le débat parlementaire. Disons-le clairement : nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux énoncés par l'intitulé de cette proposition de loi. Pourtant, des enjeux, il y en a, car parler du sport, c'est aussi parler de la société que nous voulons voir advenir, de la manière dont on se comporte avec les autres, des valeurs que l'on partage, de sa santé, de la manière dont on se déplace, dont on vit Parler du sport, c'est aussi parler de l'environnement dans lequel on le pratique, du partage de l'espace public et des équipements. Parler du sport, c'est enfin parler de celles et de ceux qui le font vivre, de leurs conditions de travail, de bénévolat et de la place de l'éducation dans ce processus. Mais de tout cela, nous ne parlerons pas aujourd'hui. Pas un mot pour répondre à la colère des professeurs d'éducation physique et sportive (EPS), qui appellent à une revalorisation de leur statut et à une autre approche du sport à l'école. Surtout, un grand vide, voire un grand déni, sur la pratique sportive de demain

et tous. On ne pratique pas le sport de la même manière quand il fait 20 degrés ou 45 degrés. Comment organiser des matchs de football en extérieur quand il fait 40 degrés à l'ombre et que la pratique sportive est déconseillée au-dessus de 32 degrés ? Non, nous ne défendons pas la solution qatarie, qui consiste à climatiser les stades ... Comment assurer l'avenir des sports d'hiver face à la fonte des glaciers et à l'absence de neige à des altitudes de plus en plus hautes ? Comment pérenniser la pratique du sport en intérieur alors que la majorité de nos gymnases ont été construits avant les années 1990 et sont des passoires thermiques ? Il n'y a là rien d'anecdotique, et beaucoup de sportifs du quotidien, tout comme des sportifs de haut niveau, nous appellent à la mobilisation générale sur ces sujets. Nous proposerons toute une série d'amendements afin que la réduction des impacts environnementaux et la résilience face aux dérèglements climatiques soient inscrites au coeur de nos politiques sportives. Parce qu'il n'y a pas de démocratisation sans inclusion, nous proposerons également le rétablissement du texte de l'Assemblée nationale pour toutes les mesures allant dans le sens de l'égalité, de l'inclusivité et de l'émancipation par le sport. Nous proposerons un certain nombre d'amendements afin que les mesures répressives à l'encontre des supporters soient justes, proportionnées et correspondent aux travaux récents des différents acteurs. acteurs. Bref, émancipation, égalité et avenir soutenable : voilà les axes de travail que nous proposerons durant nos débats. Quant à notre vote final, il dépendra du sort qui sera réservé à nos amendements, ainsi que de l'ambition que nous aurons peut-être réussi à insuffler à ce texte. La parole

à l'examen de la proposition de loi qui nous rassemble aujourd'hui, la déception prédomine : il ne s'agit malheureusement pas d'un grand texte, susceptible de régler les problèmes profonds affectant le monde du sport, en particulier du fait de la crise sanitaire. Après l'intervention de mon ami Jean-Jacques Lozach, souhaite évoquer quelques enjeux de ce texte qui me préoccupent tout particulièrement. Tout d'abord, il est question, à l'article 5, de parité au sein des fédérations agréées. Les femmes sont absentes ou extrêmement sous-représentées dans ces instances, et nombre de fédérations se plaignent des nouvelles dispositions, rigides et peu adaptées aux réalités. C'est toujours le même discours qu'on nous ressort, lorsque l'on veut s'opposer à la parité, en politique, dans les entreprises et maintenant dans le sport ! Je ne puis donc que regretter la réécriture faite en commission par notre rapporteur, qui atténue la mise en place de ce rééquilibrage par l'instauration de délais, concourant à un affaiblissement de la nécessaire obligation de parité. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présentera donc un amendement à cet article 5, fixant des objectifs de parité ambitieux, nécessaires pour les fédérations, et applicables dès le prochain renouvellement des instances. En termes de parité, un autre mauvais signal est la suppression en commission de l'article 5 A, qui prévoyait l'obligation de parité au sein du bureau du Comité national olympique et sportif français. Nous présenterons donc un amendement visant à rétablir cette obligation.

! Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s'est attaché à ce que la balance entre droits et devoirs des supporters soit équilibrée. Plusieurs amendements ont été déposés en ce sens. Ils visent à l'ouverture du capital des clubs aux supporters, au resserrement des motifs d'interdiction administrative de stade dès lors qu'une personne constitue une menace grave pour l'ordre public, ou à l'extension aux comportements homophobes de la définition du délit réprimé d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Ils tendent également à instaurer une peine d'amende pour l'introduction, la détention ou l'utilisation par les supporters, sans l'autorisation des clubs, de pyrotechnie dans les stades. Je note d'autres apports du Sénat concernant les supporters, comme l'introduction dans le texte de la possibilité d'utiliser des scanners corporels lors des manifestations sportives, même si nous trouvons que ce dispositif mériterait d'être mieux encadré. autre initiative du Sénat, la communication par la préfecture des photographies des personnes interdites de stade, dans le but de renforcer le contrôle à l'entrée des enceintes sportives, en espérant que cette disposition améliore réellement les contrôles qui sont à l'heure actuelle particulièrement chaotiques.

Un Français sur deux déclare pratiquer un sport, mais cela reste largement insuffisant, et la France se classe seulement à la dix-septième position au niveau européen en matière de pratique sportive. Le sport est une question qui touche à la santé publique, à l'éducation, à la citoyenneté. Il participe à la cohésion sociale et au rayonnement de la France, et je tiens à saluer nos athlètes qui participeront aux prochains jeux Olympiques. Le sport irrigue toute la société. Pourtant, nos politiques publiques peinent encore à refléter cette réalité. Le constat est unanime : il faut faire mieux. C'est probablement ce qui a conduit le Président de la République à dire en 2017 qu'il voulait tout mettre en oeuvre pour que la France soit une vraie nation sportive : noble cause Malheureusement, il ne s'est souvenu de son souhait que quatre ans plus tard, les jeux Olympiques de 2024 approchant à grands pas, et une pandémie étant entre-temps venue largement fragiliser l'écosystème du sport français. aujourd'hui une proposition de loi visant à démocratiser le sport, déposée par les députés de la majorité. Cette proposition s'inscrirait dans la continuité de la politique sportive de l'exécutif- mais y en a-t-il eu une ? ? Force est de constater que le plan de relance pour le sport n'est pas à la hauteur des attentes du monde sportif. Et nous attendons toujours de voir cette grande loi sur le sport et la société qui a été promise à de multiples reprises

Sans l'action de la commission de la culture du Sénat et de son rapporteur, Michel Savin, dont je salue les travaux, les questions relatives à l'EPS ou à l'engagement sportif à l'université n'auraient même pas été abordées. Rien non plus pour favoriser l'engagement associatif, souvent vieillissant, qui est pourtant la colonne vertébrale de notre modèle sportif. Rien pour soutenir les clubs face aux difficultés financières que la crise leur a causées. Rien sur la reconversion des sportifs. Rien sur le financement par l'assurance maladie de l'APA. Notons en outre que, du fait de l'examen tardif de la proposition de loi, une grande partie des dispositions en matière de gouvernance des fédérations n'auront pas d'effet avant les jeux Olympiques de 2024. Certes, je me réjouis évidemment des avancées prévues dans le texte. Je pense en particulier aux dispositions concernant l'accès aux équipements sportifs, l'honorabilité des encadrants, la lutte contre les manipulations des compétitions et contre le illégal ou encore la possibilité pour les sociétés sportives de prendre la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif.

Ce texte aurait dû être l'occasion de réinventer, sinon de renforcer notre modèle. Il aurait pu être l'occasion d'innover, par exemple en prévoyant la possibilité pour les fédérations dépourvues de ligue professionnelle de créer des ligues semi-professionnelles. Une telle mesure permettrait aux clubs amateurs évoluant à haut niveau de bénéficier d'une reconnaissance et de diversifier leurs financements.

la proposition de loi que nous examinons est le seul texte relatif au sport de tout le quinquennat. À l'approche des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris, on ne peut que regretter un tel manque d'ambition et l'absence de loi Sport et société pendant cinq ans. C'est assez décevant quand on sait que l'actuel Premier ministre a présidé l'Agence nationale du sport. En tant qu'ancienne sportive de haut niveau et double championne du monde de karaté, je le déplore. L'Assemblée nationale s'est saisie du sujet sans attendre un hypothétique projet de loi. La commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat a adopté le texte après l'avoir enrichi avec soixante-sept amendements, afin de corriger les lacunes dont il souffrait. Le texte adopté est un compromis pour rassurer et conforter le mouvement le mouvement sportif. L'un des apports principaux de la proposition de loi est le développement du sport-santé. C'est une bonne nouvelle, à l'heure où nous avons pris conscience que l'activité physique renforce notre immunité et notre bien-être. L'instauration d'une pratique sportive quotidienne dans les écoles primaires pour lutter contre la sédentarité et la promotion des activités physiques et sportives dans la formation des enseignants au sein des Inspé sont d'excellentes avancées à mettre Inscrire au titre des missions d'intérêt général et d'utilité sociale l'offre d'activités physiques et sportives des établissements sociaux et médico-sociaux conforte la dynamique à l'oeuvre depuis quelques années. À titre personnel, j'aurais souhaité que l'on puisse ouvrir la prescription d'activité physique adaptée à un public plus large, comprenant les patients atteints de pathologies physiques, mais aussi psychologiques. Je félicite la commission d'avoir formalisé un socle juridique commun des maisons sport-santé. Les collectivités territoriales sont des acteurs majeurs du soutien au sport, dont la démocratisation ne doit pas s'effectuer de nouvelles contraintes qui pèseraient principalement sur ces dernières. L'État doit y prendre une plus grande part.

La commission a eu raison de garantir leur bon fonctionnement en permettant une mise en oeuvre par étapes de la parité dans leurs instances. Je termine en évoquant le modèle économique sportif. La possibilité de création d'une société commerciale par les ligues professionnelles pour gérer et négocier les droits audiovisuels est un progrès notable, dû à l'initiative du rapporteur Michel Savin. Chers collègues, vous l'aurez compris, je suis favorable aux modifications introduites par la commission. Le groupe Les Républicains souhaite que nos débats améliorent cette version pour aboutir à un texte permettant de renforcer le monde sportif. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, présente proposition de loi répond à un véritable besoin. Alors même que la France peut s'honorer de compter un si grand nombre de licenciés, des menaces sont apparues et se sont développées avec la crise sanitaire. La pandémie a révélé l'urgence d'avoir une activité physique pour se maintenir en bonne Certains publics ont été éloignés de la pratique d'une activité sportive régulière alors que le sport joue un rôle important. Le sport ne doit pas devenir un loisir ou une activité d'initiés, ce qui peut être une pente fatale. Cela rend d'autant plus nécessaire le texte dont nous débattons. Le sport participe d'un grand nombre de principes et d'exigences : cohésion sociale, goût de l'effort, loyauté, dépassement de soi, etc. Dans ses différents rôles, je voudrais souligner un aspect traité dans le texte. « Le sport, c'est la santé » ne peut plus être qu'un simple adage. Ce doit être une véritable option, appelée à se développer et que le législateur commence à consolider. Le sport peut en effet être considéré comme une thérapie, évidemment sur le plan physique, mais aussi, et peut-être surtout, sur le plan psychique. Il contribue à l'estime de soi et à la reconstruction personnelle. Thérapie du corps, c'est aussi un soin de l'âme. Il est donc appelé à devenir un véritable traitement. C'est cette perspective qu'il faut encourager et accompagner. Mais cela suppose la prise en compte de différents paramètres. Nous saluons l'élargissement par l'Assemblée nationale du droit de prescription de l'activité physique adaptée à tout médecin, ainsi que celui du champ des bénéficiaires. La prescription d'une activité physique régulière aux personnes atteintes de maladie chronique et présentant des facteurs de risque constitue une évolution positive. Elle permet à une nécessité, la santé, et à une passion, le sport, de se rencontrer, dans une fructueuse complémentarité. Cependant, nous déplorons l'absence de prise en charge par l'assurance maladie. C'est une évolution nécessaire si l'on veut reconnaître le sport comme un véritable traitement. Le volet financier doit donc être abordé sans peur et sans pudeur. Je n'oublie pas- le problème se pose dans mon département -la faiblesse des prescriptions de sport-santé par les médecins. Est-ce le fait d'un manque d'information ou une contrainte de la part de l'assurance maladie ? Mais, en réalité, la question n'est pas tant celle du financement que celle de l'efficacité des aides et des soutiens. C'est plutôt un problème de déploiement. La complainte du manque de moyens est trop facile. Il est anormal que les publics visés ne soient pas touchés par des interventions quand ils sont censés être les premiers concernés. Il est également anormal que le sport-santé devienne une tentation lucrative ne profitant qu'à certains organismes, et non pas au grand public. Il y a évidemment un problème de communication, mais surtout une difficulté à atteindre les bénéficiaires. Il y a donc tout un travail de clarté et de transparence à poursuivre si nous voulons que le sport-santé se développe efficacement. de la plateforme en ligne recensant les offres d'APS et d'APA On constate également une carence dans la formation des cadres techniques dans les clubs pour qu'ils puissent intervenir dans le sport-santé, mais également de grosses inégalités entre les fédérations, dont les moyens sont différents. Madame la ministre, comment les pouvoirs publics agiront-ils pour que les moyens engagés atteignent réellement leur cible ? Enfin, dans ce grand effort, il faut également s'interroger sur l'apport des collectivités locales, qui seront sollicitées et mises à contribution. Cela ne pourra qu'entraîner des charges financières supplémentaires. La crainte exprimée dans le rapport de la commission de la culture est celle d'une inégalité entre les collectivités locales. Les maisons sport-santé voient leur existence formalisée par la loi, ce qui est également une avancée. Mais, sur ce plan, il faut encore envisager des implications financières pour les collectivités locales. Madame la ministre, il faut tout faire pour que les collectivités locales ne soient pas étranglées financièrement ni victimes d'une bonne idée dont elles risquent de pâtir. Il faut également faire la différence dans la distribution des moyens entre le sport adapté, le handisport et le sport-santé. En effet, dans beaucoup de départements, cela reste malheureusement une enveloppe globale et peu lisible. Ne serait-ce pas le moment de dresser un bilan d'étape sur cette stratégie nationale sport-santé, qui ne doit pas rester qu'une ambition ? La discussion

le Nord. Alors que les assemblées générales budgétaires se profilent, ces clubs n'ont toujours pas perçu la compensation prévue, qui est pourtant nécessaire à leur équilibre. Madame la ministre, auriez-vous des informations sur la date à laquelle ces associations peuvent espérer recevoir leur versement ? Quel

d'échange de bonnes pratiques et de mutualisation d'expériences, pas simplement dans un établissement précis, mais sur l'ensemble d'un territoire. En plus, cela contribue à la démocratisation des pratiques,

Oui, la pratique d'une activité sportive est vectrice de lutte contre de nombreuses pathologies, favorise le bien-être et nourrit la cohésion sociale ! Mais le fait de ne pas associer ces déclarations d'intention à de solides garanties financières les rendra vaines. avec le présent article 1, qui adosse le développement de l'activité physique à un secteur médico-social pourtant à bout de souffle. J'en profite néanmoins pour saluer le travail remarquable de Michel Savin, notre rapporteur, et de la commission, qui ont adapté ce texte à l'absence de volet financier et l'ont enrichi, insistant par exemple sur la nécessaire pratique du sport dans les écoles primaires. Loin d'être le grand projet de loi Sport et société annoncé maintes fois par l'ancienne ministre, Laura Flessel, ce texte n'est pas à la hauteur des attentes. Il oublie des acteurs essentiels, comme les associations sportives locales et leurs milliers de bénévoles, qui sont indispensables à la pratique sportive du plus grand nombre dans nos territoires. Je veux ici leur rendre hommage. aujourd'hui en grande difficulté, parfois menacées de disparition, sont la clé de l'inclusion des publics les plus éloignés des activités sportives. Elles ont été fragilisées par la suppression aveugle, dogmatique et, surtout, imbécile de la réserve parlementaire, dont personne n'a parlé. Les petits clubs locaux de village ou de quartier, qui incarnent vraiment la démocratisation du sport, ne disent pas merci au Gouvernement Ce texte, s'il a le mérite d'exister et de comporter quelques avancées, demeure à l'image de l'action gouvernementale en matière de démocratisation du sport : timide, technocratique, lacunaire et, surtout, pétri de contradictions.

Ouvrir les portes de tous ces centres aux associations sportives de territoire pour leur permettre d'intervenir et d'avoir une action beaucoup plus forte vis-à-vis de ces publics, c'est aussi les positionner différemment dans la société. Certes, la proposition de loi arrive en fin de mandat.

de la prescription médicale d'APA. Je tiens tout d'abord à rappeler que la prescription médicale d'APA au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique a une visée thérapeutique, et non préventive. Elle s'adresse aujourd'hui aux personnes souffrant d'une affection de longue durée, soit environ 10 millions d'individus. L'article 1 dans la rédaction issue des travaux de la commission étend le dispositif aux personnes atteintes de maladies chroniques, soit environ 15 millions de personnes supplémentaires. Cela ferait donc une population totale de 25 millions de personnes.

déficit de formation des médecins, notamment s'agissant de l'orientation vers l'APA ; problèmes d'accessibilité géographique de l'offre. Avec l'ouverture du dispositif à de nombreux bénéficiaires, l'enjeu réside désormais dans la capacité du système à répondre à la demande et à garantir l'effectivité de l'APA.

effet, pour la majorité des personnes concernées, c'est la parole d'un professionnel de santé qui est crédible et légitime. Nous avons signé avec l'ordre des médecins une convention par laquelle ils s'engagent à répandre la bonne parole, à former, à convaincre encore

Si le Président de la République a inscrit dans ses engagements la labellisation de 500 maisons sport-santé, c'est parce qu'il faut en priorité faciliter la structuration de ces acteurs. Aujourd'hui, nous en comptons 436, en incluant la dernière que j'ai visitée, près de Limours.

en réécrivant l'article et en supprimant la limitation aux affections de longue durée. En effet, de nombreuses maladies, non reconnues comme des maladies chroniques ou des affections de longue durée, nécessitent pourtant un parcours de soins qui pourrait inclure l'activité physique adaptée. C'est par exemple le cas du covid long, qui pourrait bénéficier de la prescription d'une activité physique adaptée comme soin de réadaptation et de rééducation. L'enquête réalisée par Santé publique France dans le cadre de la crise sanitaire, publiée le 4 février 2021, le 4 février 2021, témoigne, à l'instar de nombreuses études scientifiques, des liens étroits existant entre troubles anxieux et dépressifs, insuffisance d'activité physique et comportements sédentaires. La parole

proposons ainsi d'ouvrir la prescription du sport-santé à un public plus large, comprenant les patients atteints de pathologies physiques et psychologiques. Bien que de nombreuses maladies ne soient pas reconnues comme des maladies chroniques ou des affections de longue durée, des patients peuvent avoir besoin d'une prescription d'activité physique adaptée, en accord avec leur médecin. C'est le cas des personnes atteintes de dépression. Sans qu'elle constitue un remède miracle, il est reconnu que l'activité physique est un moyen concourant à soigner les troubles anxieux, les troubles psychiques les dépressions, en complément ou en remplacement de médicaments spécifiques. L'expérience des confinements depuis le début de la crise sanitaire a encore renforcé cette prise de conscience, en mettant en avant un lien évident entre les dépressions et le manque d'activité physique et la sédentarité. Je suis heureuse d'entendre que des projets de remboursement par la sécurité sociale sont envisagés. Je regrette simplement qu'ils arrivent en fin de quinquennat ... L'amendement

est à M. Éric Gold. Par cet amendement, je souhaite, à l'instar de mes collègues, souligner l'intérêt du dispositif de l'activité physique adaptée. Comme je l'ai rappelé lors de la discussion générale, les gains pour la santé physique et psychologique sont immenses et les coûts évités le sont tout autant. Le sport est un véritable médicament. L'étude de l'Inserm réalisée en 2019 à la demande du Gouvernement l'illustre clairement et recommande fortement cette prescription pour de nombreuses pathologies. Aussi, élargir cette prescription comme le fait le texte aux patients atteints de maladies chroniques ou présentant des facteurs de risque tels que le surpoids, l'obésité

Florence Lassarade, pour présenter l'amendement n° 36 rectifié Cet amendement vise à permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de prescrire une activité physique adaptée aux patients atteints d'une affection de longue durée. Cette mesure permettra de lever les freins sur le développement de ce dispositif dont l'efficacité n'est plus à prouver en matière de santé publique. Les kinésithérapeutes sont en effet des professionnels de santé, mais des professionnels du sport, qui, dans leurs activités de soin et de prévention, utilisent l'activité physique et sportive. Dans son rapport sur la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, la Cour des comptes soulignait « l'échec de la prescription médicale d'activité physique adaptée », considérant que cet échec était notamment imputable à la « restriction de la prescription aux seuls médecins traitants, alors que des médecins spécialistes sont très mobilisés sur le sujet » et à une « présentation par profil de limitations fonctionnelles complexe à appréhender pour les médecins généralistes non formés ». La mise en oeuvre d'une activité physique adaptée ne peut être soumise à prescription obligatoire. En effet, il s'agit d'une action de prévention dispensée au moyen de techniques physiques et sportives, et non d'un acte thérapeutique. Dès lors, l'élargissement de la possibilité de prescription de l'APA aux masseurs-kinésithérapeutes a pour objectif de promouvoir cette activité auprès des patients. Élargir la possibilité de prescrire une activité physique adaptée aux masseurs-kinésithérapeutes permettrait de répondre à ce manque de relais et de développer davantage ces pratiques. D'autre part, un nombre croissant de nos concitoyens rencontrent des difficultés pour accéder aux soins : 10 % n'ont plus de médecin traitant. Un droit de prescription élargi à l'APA permettrait de libérer du temps médical, d'éviter certains déplacements superflus et d'améliorer l'efficience de l'équipe de soins en mettant à profit les compétences des médecins spécialistes- rhumatologue, oncologue, cardiologue ... -et des masseurs-kinésithérapeutes. De plus, les masseurs-kinésithérapeutes sont déjà au contact des patients porteurs d'une ALD susceptibles de bénéficier de ce dispositif. Interlocuteurs de proximité, ils suivent ces patients dans leur parcours de soins de façon souvent hebdomadaire et sont les seuls professionnels de santé à être également des professionnels du sport du sport selon l'article A. 212-1 du code du sport. Les masseurs-kinésithérapeutes sont en effet les professionnels de santé spécialistes de la rééducation fonctionnelle et motrice et de la réadaptation. Ils utilisent à cette fin l'activité physique et sportive. Enfin, le recours à un professionnel de santé s'avère indispensable pour intégrer réellement l'activité physique dans le parcours de soins en offrant aux patients un véritable cadre thérapeutique et en assurant leur prise en charge dans le respect de leurs droits fondamentaux, tels que le secret professionnel.

Je connais la réponse du rapporteur et la position de la commission, favorable au renouvellement, défavorable à la prescription. Toutefois, limiter à certaines professions et à certains professionnels de santé la prescription, c'est écarter de fait un grand nombre de patients

L'ouverture du droit de prescription de l'APA, aujourd'hui limité aux seuls médecins traitants, est effectivement l'un des leviers à son déploiement à une plus large échelle. En étendant ce droit à tous les médecins intervenant dans la prise en charge des patients, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, l'article 1 constitue une avancée importante. Il m'a semblé qu'une étape supplémentaire pouvait être franchie en permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de renouveler et d'adapter

plus loin, en autorisant les masseurs-kinésithérapeutes à prescrire l'APA. J'y suis défavorable pour deux raisons. Premièrement, la prescription d'APA concerne actuellement des patients souffrant d'une affection de longue durée, et bientôt ceux atteints d'une maladie chronique figurant sur une liste déterminée par décret, si le présent texte est adopté. On parle donc bien de personnes ayant une pathologie. Dès lors, un avis médical initial me semble indispensable : les médecins intervenant dans la prise en charge de ces personnes sont en effet ceux qui connaissent le mieux leur maladie et qui sont les plus aptes à juger de la pertinence d'une prescription d'APA et de ses modalités. Deuxièmement, le droit pour les masseurs-kinésithérapeutes de renouveler et d'adapter les prescriptions médicales d'actes de masso-kinésithérapie n'est devenu effectif que depuis 2021. J'ai souhaité que cette possibilité très récente soit étendue aux primo-prescriptions médicales d'APA. Ces deux dispositifs constituent déjà des avancées majeures pour les masseurs-kinésithérapeutes.

M. Stéphane Piednoir. Cet amendement vise à prendre en compte les activités physiques et sportives dans les négociations professionnelles annuelles. L'article L. 4121-1 du code du travail confie à l'employeur le soin de protéger la santé des travailleurs.

Sénat, l'exclusion de l'assiette sociale des avantages relatifs à la pratique du sport en entreprise, jusqu'alors encadrés par voie réglementaire. Cette mesure, très attendue, a été déclinée dans le décret du 28 mai 2021 relatif aux avantages liés à la pratique du sport en entreprise.

a permis aux entreprises d'inscrire dans leurs statuts une raison d'être, à savoir une ambition d'intérêt général qu'elles entendent poursuivre dans le cadre de leur activité. Le sport, au travers de sa force de développement individuel,

en considération, au même titre que les enjeux sociétaux et environnementaux, par le conseil d'administration ou le directoire d'une société au moment de déterminer les orientations de son activité. Cette disposition participe pleinement

la présence d'un référent sport au sein des maisons départementales des personnes handicapées, qui font souvent office de guichet quasi unique pour les personnes en situation de handicap dans les territoires. Ce sont vers elles que se tournent ces personnes pour nombre de démarches, y compris celles relatives au sport

rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale faisait une claire mention de l'intégration sociale, de la solidarité intergénérationnelle et de la vie démocratique. L'accent était également mis sur l'égalité des chances, sur la préservation de la santé, du bien-être moral et physique des individus et, plus généralement, sur l'épanouissement de la personne et le progrès collectif.

sportives font partie intégrante de l'éducation et de la culture et permettent l'apprentissage de la citoyenneté, de la solidarité entre les générations et de l'intégration

au deuxième alinéa, l'apprentissage des principes et des valeurs de la République. Ces dernières sont écrites au fronton de toutes les mairies : liberté, égalité, fraternité, auxquelles certains ajoutent parfois la laïcité, même si cela fait débat. Les principes de la République, eux, sont énoncés

pas synonymes de dangerosité. Si le sport se doit d'être émancipateur pour les individus, ne jetons pas l'opprobre sur celles et ceux qui le pratiquent dans le respect de leurs croyances. Il faut d'urgence pacifier ce débat et s'interroger sur ce contre quoi nous voulons lutter. Le combat quotidien contre toutes les formes de radicalisation doit être au coeur de nos principes, mais il doit

Cet amendement vise à supprimer la référence particulière à la laïcité, introduite en commission, au motif qu'elle fait déjà partie des principes de la République.

Pourtant, les études ont très largement démontré que ceux qui souffrent d'anxiété, de troubles bipolaires ou encore de schizophrénie sont majoritairement des personnes qui ne se dépensent pas physiquement de façon régulière.

contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. » Il ajoute également que « L'État et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales,

ensemble, non pour travailler à leurs côtés ou à leur place. J'en profite pour saluer le travail de l'Agence et des agents de mon ministère, qui déploient sur les territoires une partie des dispositifs que l'ANS a pour mission de financer ou de cofinancer.

Cet article vise à reconnaître le rôle de l'Agence nationale du sport, qui a été créée pour mettre en oeuvre une gouvernance partagée

et déterminer les choix d'investissement dans les territoires. L'ANS est ainsi l'instance qui débat sur les demandes de participation financière des collectivités, soit au niveau national, soit au niveau des conférences régionales.

et des spectateurs. Le bilan carbone est loin d'être négligeable. En optimisant les déplacements, on peut réduire non seulement les émissions de CO2, mais aussi la fatigue induite pour les participants. Vingt-huit fédérations sportives utilisent aujourd'hui un logiciel d'optimisation des rencontres sportives au regard du nombre de kilomètres réalisés, appelé

Pourtant, le sport, qui est obligatoire tout au long de la scolarité des élèves, disparaît complètement lorsque les jeunes quittent le lycée et entrent dans l'enseignement supérieur. Les étudiants ne sont plus incités à pratiquer une activité physique sportive régulière, quasi quotidienne, comme ils ont pu l'être durant leur scolarité primaire et secondaire. L'objectif des auteurs de cet amendement est

Selon les chiffres d'une étude de l'IFOP, en janvier 2021, 27 % des enseignants d'éducation physique et sportive disent avoir déjà observé une forme de contestation de l'enseignement par un élève au nom de la religion. C'est tout à fait comparable avec les pourcentages que l'on observe pour les enseignements abordant la laïcité- 26 % - ou pour les enseignements abordant l'éducation à la sexualité ou l'égalité filles-garçons, à hauteur de 25 %. Par ailleurs, 40 % des enseignants disent avoir déjà observé des absences de jeunes filles à des cours d'EPS au nom de convictions religieuses, avec ou sans certificat médical.

fait partie des enseignements obligatoires et que la non-participation aux activités sportives ne peut reposer que sur des raisons médicales. Cet amendement vise donc à lutter contre les certificats médicaux de complaisance et à créer une alerte à chaque fois que le motif réel de l'inaptitude de l'élève est mis en doute.

Au même titre que les autres enseignements, l'EPS est obligatoire. En cas d'inaptitude totale ou partielle, il faut justifier d'un certificat médical, qui doit préciser le type d'inaptitude au regard d'un type de mouvement, d'effort, de durée et d'environnement. un enfant vient avec un tel certificat, on peut toujours lui proposer d'adapter la pratique physique et sportive pour la rendre compatible avec son inaptitude. En cas de certificat de plus de trois mois, une visite du médecin scolaire peut être proposée à l'élève. Dans tous les cas, si les précisions du médecin ayant délivré le certificat sont jugées insuffisantes, le médecin de l'éducation nationale peut être sollicité, quelle que soit la durée de validité du certificat, notamment s'il est supérieur à trois mois. De mon point de vue, il n'y a pas lieu de renforcer le contrôle des médecins scolaires sur ces certificats médicaux

principes de la République. Chacun peut exercer librement sa religion, mais, sur un terrain de sport, la neutralité doit s'imposer. Il me paraît essentiel qu'il n'y ait pas de différence ou d'appartenance particulière à mettre en avant sur un terrain de sport, de quelque nature qu'il soit. Aujourd'hui, un flou juridique existe sur le port de signes religieux. Il est nécessaire que l'État définisse clairement les règles. Si le port du voile n'est pas explicitement interdit, on pourrait voir émerger des clubs sportifs communautaires promouvant certains signes religieux.

une généralité. Cet amendement vise donc à clarifier la situation et à demander à l'État de prendre ses responsabilités pour imposer la neutralité sur tous les terrains de sport, quels qu'ils soient.

lors des compétitions sportives. Certaines fédérations les interdisent, d'autres les autorisent. Ces divergences sont peu compréhensibles pour les pratiquants. Un contentieux est d'ailleurs en cours devant le Conseil d'État sur le droit d'une fédération sportive d'interdire tout discours ou affichage pour le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. En l'occurrence, c'est de la Fédération française de football qu'il s'agit, un collectif de « hidjabeuses » ayant remis en question le règlement fédéral,

républicain commun repose notamment sur le principe de laïcité, qui garantit à la fois la neutralité de l'État à l'égard de tous les cultes et la liberté de croyance religieuse de nos concitoyens.

Le Gouvernement s'est pleinement engagé sur le sujet du séparatisme depuis le début du quinquennat. Le nouveau contrat d'engagement républicain, mis en place par la loi d'août 2021 confortant le respect des principes de la République, engage désormais expressément les associations sportives et les fédérations

en tenant compte, notamment, des objectifs liés à l'ordre public et au bon fonctionnement des associations. Ce contrat d'engagement républicain est désormais obligatoire. Le décret d'application a été publié le 1 janvier dernier. Il comporte l'engagement, pour les associations et les fédérations sportives, de s'abstenir de tout acte de prosélytisme abusif, exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression.

en augmentation à travers les conventions conclues par l'Agence nationale du sport. Cette dernière doit, elle aussi, se doter d'une charte relative aux valeurs de la République pour encadrer son action.

de promotion du carré régalien du sport : lutter contre les séparatismes, prévenir les violences et les discriminations, améliorer le fonctionnement démocratique et prendre en compte les enjeux environnementaux. est la RSE du sport sur laquelle le Gouvernement s'engage. La lutte contre le séparatisme et les dérives communautaire en fait pleinement partie. Toutes les fédérations délégataires, qui reçoivent une mission et un monopole de la part de l'État, seront tenues de s'engager et de contrôler activement leurs associations.

travaillerons encore davantage de concert pour former nos éducateurs sportifs, ainsi que nos professeurs des écoles, à cette thématique : il importe qu'ils sachent comment l'appréhender. Depuis ma prise de fonction, j'ai organisé plusieurs séminaires de deux jours avec tous ces réseaux.

mobilisation, coordination, sensibilisation, coopération, contrat et pacte. Ce n'est

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Merci,

mais aussi les ceux inscrits sur la liste des sportifs espoirs, sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ou des centres de formation d'un club professionnel.

déjà mise en oeuvre. Pourtant, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 612-3 du code de l'éducation ne fait mention que des sportifs de haut niveau, dont la liste est mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport.

publique faisant l'objet d'une réhabilitation peut parfois s'avérer impossible en raison de contraintes foncières ou de règles urbanistiques. Le travail en commission a permis de prendre en compte cette situation d'un point de vue financier.

par de nombreux sportifs. Il s'agit aussi d'une forme de reconnaissance de l'action et de l'investissement des collectivités locales dans le cadre du développement des activités de proximité pour aménager les espaces publics, notamment avec des équipements sportifs, des jardins publics et autres parcs. Avis favorable.

2 de la proposition de loi prévoit un recensement par académie des locaux et équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement physique et sportif. Cette mesure est bienvenue. Nous proposons de l'améliorer en prévoyant que le recensement prenne en compte les performances énergétiques des équipements et leur résilience face aux dérèglements climatiques. Toutes les activités humaines ont un impact sur l'environnement ; le sport ne fait pas exception. Les gymnases, piscines et salles de sport sont consommatrices d'énergie, notamment par l'éclairage et le chauffage des bâtiments. Il apparaît ainsi indispensable que les services de l'État connaissent la performance énergétique de ces équipements pour réduire leur empreinte, particulièrement après les annonces sur les 5 000 équipements bénéficiant du plan de relance. Par ailleurs, nous le savons, quelle que soit la trajectoire que l'humanité va emprunter pour réduire ses émissions, le dérèglement climatique est une réalité qui commence déjà à produire des effets dramatiques, avec des des intempéries de plus en plus fréquentes, des canicules et des pics de chaleur généralisés et de plus en plus longs. La pratique sportive s'en trouvera nécessairement bouleversée. Selon WWF, dans un scénario de dérèglement climatique et d'une hausse des températures de 4 degrés, les Français pourraient perdre jusqu'à deux mois d'activité sportive

l'amendement n° 66. À l'Assemblée nationale, une disposition intéressante avait été introduite en commission : l'obligation faite aux établissements scolaires privés, dès lors qu'ils reçoivent une subvention publique, de mettre à la disposition des établissements scolaires publics

puisqu'il est spécifiquement précisé que la mutualisation a lieu pendant les heures ou les périodes au cours desquelles lesdits équipements ne sont pas utilisés. Enfin, l'enseignement privé a été suffisamment avantagé par la présente proposition de loi, un amendement de notre rapporteur les ayant retirés de l'obligation prévue à l'article 2 de créer un accès indépendant à leurs équipements sportifs.

Il remet en cause implicitement le principe de la participation financière publique à l'école privée sous contrat. Il pose un problème d'immixtion du législateur dans la fixation du prix par une personne privée. Enfin, la personne publique bénéficiaire d'une mise à disposition à un tarif plus avantageux n'est pas forcément celle qui a accordé la subvention, ce qui peut également poser des problèmes entre collectivités : certaines vont apporter des subventions et d'autres vont bénéficier

monsieur le rapporteur.

Cet amendement vise à supprimer la mention de la neutralité des locaux publics utilisés pour le sport en dehors du temps scolaire. J'ai eu longuement l'occasion de m'exprimer sur l'engagement du Gouvernement en matière de lutte contre le séparatisme religieux et les dérives communautaires. évoqué les nouvelles obligations qui vont incomber aux associations sportives et aux fédérations sportives pour lutter contre le prosélytisme abusif. Je voudrais rappeler que, selon la Constitution, le principe de neutralité n'est pas applicable lors de l'utilisation de locaux publics pour la pratique sportive, sauf lorsqu'il s'agit de sport relevant du temps scolaire. En effet, les usagers de ces locaux hors du temps scolaire ne sont pas soumis au respect du principe de neutralité, puisque seuls les élèves le sont, ainsi que les salariés des associations qui exercent une mission de service public pour les fédérations délégataires.

Ces bons, qui permettraient de payer tout ou partie d'une licence ou d'une adhésion à une association sportive ou à un club sportif, seraient proposés par l'employeur aux salariés, dans des conditions fixées par décret. Cette disposition s'inscrit pleinement dans l'esprit de la présente proposition de loi de démocratiser la pratique sportive et de développer le sport-santé. Favoriser la pratique du sport au sein de la population active contribue à limiter les risques liés à la sédentarité et améliore l'état de santé de nos salariés.

de la déclinaison territoriale de la nouvelle gouvernance du sport, et notamment de l'ANS. Ils sont sans doute indispensables pour alimenter le travail et le contenu

M. Thomas Dossus. Les plans sportifs locaux vont permettre de réunir les acteurs de terrain et les collectivités pour développer la pratique sportive dans les territoires. La méthode et l'objectif nous semblent bons,

y associer les usagers du sport, car tous les sportifs ne sont pas licenciés ou n'appartiennent pas au mouvement sportif en tant que tel. Les citoyennes et citoyens pratiquant le sport, quel que soit leur niveau d'implication, doivent pouvoir être démocratiquement associés aux plans locaux. Nous sommes bien au coeur de l'objectif de cette loi : la démocratisation du sport. Quel

Lozach. Cet amendement vise à faire valider les plans sportifs locaux par un conseil local des APS, dont la composition et les modalités seraient déterminées par décret. Quel est l'avis de

actuellement concourir au développement des associations sportives scolaires du premier degré. La nouvelle rédaction de l'article L. 552-2 du code de l'éducation proposée par le Gouvernement mentionnerait uniquement les collectivités participant à un plan sportif local. sportif local. Les communes et groupements de communes n'ayant pas de plan sportif local, tout comme les départements et les régions, ne seraient plus incités à concourir au développement de ces associations. Enfin, la notion d'alliance éducative territoriale nous paraît floue.

n'allons pas nous laisser bercer avec des paroles. M. Jean-Michel Blanquer nous a déjà fait le coup sur un sujet que je connais intimement, qui s'appelle la Rentrée en musique.

Les associations sont exsangues ; elles ont du mal à redémarrer après l'épisode du covid. Si vous voulez du sport et de la musique à l'école

local (DSIL). Le sport intervenant de façon transversale sur les différentes catégories d'opérations prioritaires, qu'il s'agisse de la transition énergétique, de la réalisation d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement de la population, de la mise aux normes et de la sécurisation des équipements publics,

Génération 2024 » auprès des écoles. Or, lorsqu'une école veut être labellisée « Génération 2024 », elle a l'obligation d'avoir une association sportive.

M. Thomas Dossus. Nous souhaitons que les comités régionaux, territoriaux et départementaux olympiques et sportifs puissent être associés, à leur demande et selon l'échelle géographique pertinente,

Nous sommes persuadés que l'aménagement du territoire est un outil puissant de développement de la pratique sportive ; encore faut-il que des principes clairs soient énoncés dans la loi. Nous proposons ici d'inclure le développement des activités physiques et sportives dans les orientations des documents d'urbanisme, SCoT et PLUi. Nous souhaitons également que la promotion des activités sportives soit inscrite dans les principes généraux de l'action des collectivités en matière d'urbanisme. La promotion généralisée des activités physiques et sportives a un impact plus que bénéfique sur la santé des citoyens, toutes les études le démontrent. Mais elle

dans le cadre du projet éducatif territorial, lequel permet l'organisation d'activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation. Il s'agit toujours de donner corps à l'idée de parcours sportif de l'enfant

Merci,